Madame la présidente,

mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, c'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour l'examen de cette proposition de loi relative à la création du Centre national de la musique. Vous le savez, c'est un projet qui me tient à coeur depuis maintenant longtemps. Dès 2011, j'avais participé aux premières réflexions sur le sujet, aux côtés de Didier Selles, d'Alain Chamfort, de Daniel Colling et de Marc Thonon. Malheureusement, nos préconisations n'avaient pas été suivies à l'époque et les choix politiques du début du précédent quinquennat avaient conduit à mettre ce projet en sommeil. Mais aujourd'hui, nous y voilà ! Aujourd'hui, ce projet est enfin en passe d'aboutir ! L'adoption de cette proposition de loi permettra au Centre national de la musique de voir le jour, dès le 1 janvier prochain. C'est une échéance ambitieuse,

La musique, c'est d'ailleurs la première pratique culturelle des Français. Elle est l'art démocratique par excellence, un art qui permet, davantage encore que les autres, de faire tomber les barrières culturelles et sociales, parce que la musique a ceci d'universel qu'elle parle à chacun d'entre nous, parce qu'il n'y a besoin d'aucun prérequis pour être ému par une mélodie, parce qu'il n'y a pas besoin de connaître l'histoire de la musique classique pour vibrer au son du violon de Renaud Capuçon, parce qu'il n'y a pas besoin de comprendre les paroles d'Aya Nakamura pour pouvoir les chanter. La musique, c'est aussi un puissant levier de liberté, une clé pour l'émancipation, y compris dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou les zones rurales isolées. De NTM hier jusqu'à PNL aujourd'hui, combien d'artistes sont issus de ces quartiers dont on leur disait qu'ils ne pourraient jamais sortir ? De Madeon à Kungs, combien de DJ ont été révélés au grand jour en postant, depuis leur chambre, des sur SoundCloud ou YouTube ? Ils nous apportent la preuve, comme tant et tant d'autres artistes, que les professionnels de la musique de demain, ce sont les passionnés d'aujourd'hui. À ce propos, je veux rappeler l'importance des pratiques musicales amateurs. Monsieur le rapporteur, cher Jean-Raymond Hugonet, je sais que vous y êtes, comme moi, très attaché. Si le Centre national de la musique a comme vocation principale de soutenir les professionnels du secteur, il sera également au service de tous les passionnés de musique, au travers notamment de ses missions d'information. La musique, c'est, enfin, l'une des principales industries culturelles du pays, par son dynamisme économique et son rayonnement international, rayonnement dont témoigne la présence en nombre des artistes français sur les scènes des festivals de l'été du monde entier.

par l'essor du numérique, par la révolution des modes d'écoute, par la crise du disque qu'elle a subi de plein fouet, par le piratage de masse. De fait, entre 2002 et 2015, la musique enregistrée a perdu 60 % de son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, l'industrie semble avoir surmonté la crise qu'elle a eu à traverser. Depuis 2016, elle renoue avec la croissance, principalement grâce à l'essor de la diffusion en flux- le ministre chargé de la francophonie ne saurait utiliser, surtout dans cet hémicycle, un autre terme, mais vous voyez bien de quoi il s'agit ! Toutefois, il convient de rester très prudents, le secteur demeurant fragile à plusieurs égards. La diffusion en flux peut être porteuse de menaces pour la diversité musicale, avec un risque de concentration des écoutes sur quelques artistes et genres musicaux les plus populaires, renforcé par les algorithmes de recommandation des plateformes. Plus largement, la position dominante de quelques grandes plateformes peut fragiliser l'écosystème musical dans son ensemble. L'essor de ces nouveaux modes de diffusion efface les frontières et accroît la concurrence internationale. C'est une formidable opportunité pour la diffusion des artistes français à l'étranger, mais c'est aussi, potentiellement, une menace pour la place de la création musicale française et francophone dans notre pays. Le spectacle vivant musical a connu un dynamisme remarquable au cours des dernières années, malgré les attentats infâmes qu'il a eu à subir, de Paris à Manchester. Là encore, la musique a fait la preuve de son pouvoir de rassemblement et de communion. Cependant, c'est un secteur qui est, lui aussi, exposé à un risque de concentration excessive. Il a connu l'an dernier un ralentissement de son activité, dont tout le monde espère qu'il soit purement conjoncturel. Par ailleurs, la distinction entre spectacle vivant et musique enregistrée apparaît de moins en moins opérante. Les acteurs conçoivent désormais leur développement artistique et économique de manière de plus en plus intégrée, selon des stratégies dites, de façon imagée, « à 360° », qui mettent le créateur, qu'il soit auteur ou artiste-interprète, au centre du projet. Ces bouleversements profonds ont fait voler en éclat les vieux clivages. Il est temps d'en tirer les conséquences. Il est temps de rationaliser, d'adapter et de renforcer nos outils de soutien, d'accompagnement et d'observation de la filière musicale. Il est temps de les rassembler au sein d'une maison commune : c'est tout l'objet de la création du Centre national de la musique. devra être au service de l'ensemble de la filière musicale et de toutes les esthétiques. Les soutiens économiques qu'il mettra en oeuvre seront conçus de manière à promouvoir la diversité culturelle et à favoriser l'innovation. Il placera les dimensions territoriales et internationales au coeur de son action. Il viendra compléter et amplifier l'action que mènent, au quotidien, dans le domaine musical, les directions régionales des affaires culturelles de mon ministère, en lien étroit avec les collectivités territoriales. Il aura, en outre, une mission essentielle d'observation, de veille et de prospective. Les études qui seront conduites à ce titre permettront à la fois d'évaluer l'efficacité des dispositifs de soutien- je pense, notamment, aux crédits d'impôt, dont le Parlement a souhaité, lors de la discussion budgétaire, qu'ils soient mieux suivis -et d'éclairer les enjeux de partage de la valeur, d'accompagnement de la transition numérique et de promotion de la diversité musicale face aux phénomènes de concentration. Ces études pourront ainsi nourrir les réflexions sur l'amélioration de nos mécanismes de régulation, qui resteront du ressort de l'administration centrale. Afin de préparer les conditions de la mise en place du Centre national de la musique, j'ai installé, à la fin du mois de mars, un comité opérationnel. J'en ai confié la présidence à l'inspectrice générale des affaires culturelles Catherine Ruggeri. Par sa longue expérience dans le domaine culturel et musical, par sa connaissance de l'administration et par sa capacité à prendre en compte les positions de tous les acteurs, elle m'a semblé être la personne la plus à même de conduire cette mission délicate. Le comité qu'elle préside, qui se réunit toutes les semaines depuis maintenant plus d'un mois, est composé des directeurs des structures appelées à être fédérées au sein du Centre national de la musique et de représentants des services compétents du ministère de la culture, bien évidemment. En s'appuyant sur la présente proposition de loi, ce comité a pour mission de mener tous les chantiers juridiques, budgétaires, administratifs, immobiliers, informatiques et sociaux devant aboutir à la création du Centre national de la musique au début de l'année 2020. J'insiste particulièrement sur la dimension humaine du projet. Je tiens à ce qu'une attention particulière soit portée aux salariés des différents organismes appelés à intégrer le CNM, ainsi qu'aux conditions de leur transfert. Les travaux du comité avancent à un bon rythme, ce dont je me réjouis. Je suis notamment heureux de pouvoir annoncer le lancement par mes services, en lien avec le comité opérationnel et les organismes de gestion collective, de deux études économiques, l'une aux artistes, l'autre aux entreprises de la musique. Ces études constitueront un premier jalon de la fonction d'observation du secteur dévolue au CNM. Elles lui permettront également d'asseoir ses futurs régimes d'aides sur une base robuste de connaissance du marché et de ses acteurs, condition de leur efficacité. Leurs résultats devraient être connus avant la fin de l'année. J'ai souhaité également, toujours dans une logique de concertation et d'adhésion, que les acteurs et les professionnels du secteur soient pleinement associés à ces réflexions. C'est ainsi qu'un comité élargi, intégrant l'ensemble des représentants de la filière, a été créé pour échanger régulièrement avec Catherine Ruggeri et le comité opérationnel. Il s'est réuni pour la deuxième fois en juin. Je sais que les échanges ont été extrêmement riches et positifs, notamment sur la « petite loi » issue des travaux de l'Assemblée nationale. Il se réunira pour la troisième fois le 26 juillet, ce qui devrait fournir l'occasion d'évoquer le projet de décret statutaire du Centre national de la musique, qui viendra préciser les conditions d'application de la présente loi. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je vous l'ai dit et je le répète, ce projet me tient tout particulièrement à coeur, et ce depuis longtemps ! Vous pouvez compter sur moi pour mettre toute mon énergie et toute ma volonté au service de sa concrétisation. Je suis à vos côtés pour défendre la diversité de la création musicale, qui nous est si chère. Ce projet représente un nouvel élan pour la filière musicale. Cette proposition de loi, ce sont des garanties nouvelles pour ses acteurs. C'est un texte cohérent et équilibré, et je souhaite sincèrement remercier toutes celles et tous ceux avec lesquels mon ministère et moi-même avons pu mener un travail fertile

J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt vos débats. Je tiens à saluer, en particulier, plusieurs évolutions adoptées en commission, que le Gouvernement soutient pleinement. Vous avez continué, à juste titre, à élargir le champ des missions dévolues au Centre national de la musique Je pense à la pleine inclusion des variétés, y compris l'humour et le cabaret, non seulement dans le domaine du spectacle vivant, mais aussi dans celui de l'enregistrement phonographique. C'est une clarification très utile. Je suis aussi très favorable aux enrichissements que vous avez apportés aux missions du Centre national de la musique concernant la protection de l'environnement et le développement durable. C'est essentiel pour notre avenir et celui des générations futures, et ce sont des préoccupations qui doivent désormais irriguer et orienter toutes nos politiques publiques. Le renforcement des compétences du CNM en matière de collecte et de diffusion d'informations économiques et statistiques apparaît, quant à lui, pleinement cohérent avec sa dimension centrale d'observation du secteur. Enfin, la possibilité expresse qu'auront les collectivités territoriales de conclure des contrats et de nouer des partenariats avec le Centre national de la musique va dans le sens du renforcement de sa dimension territoriale.

texte aujourd'hui en séance publique devrait fournir l'occasion d'en améliorer encore la rédaction. Je pense en particulier, cher Jean-Raymond Hugonet, à l'amendement que vous avez déposé pour préciser les contours de la notion de création, sans doute trop floue et surtout liée à l'univers du spectacle vivant. Son remplacement par celles d'écriture, de composition et d'interprétation permet de renvoyer aux catégories juridiques, bien établies et chères aux organismes de gestion collective, d'auteurs, de compositeurs et d'interprètes. Le Gouvernement est donc pleinement favorable à l'adoption de cet amendement. Naturellement- vos débats en commission s'en sont fait l'écho -, le texte dont nous discutons aujourd'hui n'a pas vocation à fixer dans le détail l'ensemble des règles de fonctionnement du futur CNM. J'ai perçu, en particulier, l'intérêt bien légitime que vous portez aux questions de gouvernance et de financement. Je suis conscient que ces deux sujets sont absolument essentiels. On ne construira pas le CNM sans un effort financier à la mesure des enjeux, allant au-delà des ressources actuelles du CNV, actuelles du CNV, et sans une gouvernance permettant de concilier efficacité, agilité et association des parties prenantes au projet. Mais il y a un temps pour tout le financement du CNM sera précisé lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2020 et sa gouvernance sera définie dans le décret statutaire en cours de préparation. qui concerne le financement, j'ai entendu les craintes de certains acteurs de la filière quant à la continuité avec le système actuel. Il n'est pas souhaitable de rigidifier le fonctionnement par une politique de fléchage,

En ce qui concerne plus spécifiquement les réserves du CNV, il est essentiel qu'elles soient employées dans le cadre du périmètre actuel de l'établissement public. Quant à la gouvernance du CNM, qui sera un établissement public, elle devra être resserrée et assurer, conformément aux préconisations de la mission parlementaire, une place majoritaire à l'État au sein du conseil d'administration. L'association des représentants du secteur sera notamment garantie par la présence d'un comité professionnel. La représentation des territoires sera, quant à elle, pleinement assurée, que ce soit au conseil d'administration ou au conseil professionnel. L'amendement adopté en commission élargissant la composition du conseil professionnel aux représentants d'organisations publiques, et non plus seulement privées, va, à ce titre, dans le bon sens. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, l'union : voilà ce qui doit présider au projet de Centre national de la musique Elle a prévalu à l'Assemblée nationale, puisque la proposition de loi y a été adoptée à la quasi-unanimité. C'est le signe d'un soutien large, qui dépasse les clivages politiques. Je m'en réjouis sincèrement. Je ne doute pas que le même esprit d'union prévaudra dans cet hémicycle. C'est en confirmant aujourd'hui cette dynamique vertueuse que vous parviendrez, je l'espère, à un accord en commission mixte paritaire par la suite un accord qui ouvrira la voie à une promulgation rapide de cette belle et importante loi pour le secteur musical et, plus largement, pour la culture dans notre pays ; un accord qui ouvrira la voie à la mise en oeuvre résolue de ce beau projet. La parole

Malheureusement, en 2012, alors que l'ensemble des acteurs étaient prêts à s'engager, le projet avait été abandonné, faute de moyens ; la filière en garde un fort ressentiment. Dans ce contexte, la relance du projet du Centre national de la musique au printemps de 2017 par Françoise Nyssen, alors ministre de la culture, que je veux saluer ici, a fait renaître beaucoup d'espoirs. Les conclusions du rapport de Roch-Olivier Maistre, qui confirmaient l'intérêt de créer un établissement public chargé d'observer, d'appuyer le développement international et de soutenir le secteur dans une optique de diversité culturelle, ont été unanimement saluées par les acteurs de la filière musicale. La mission de préfiguration du CNM, confiée aux députés Pascal Bois et Émilie Cariou, a débouché sur le dépôt, le 27 mars dernier, d'une proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale le 6 mai. Monsieur le ministre, vous avez donc été l'homme à l'origine de ce projet, mais vous serez bientôt aussi l'homme à sa conclusion, qui doit constituer, nous le pensons tous ici, un nouveau départ pour le monde de la musique en France. Pourquoi est-il si important de donner corps à ce projet ? Nous avons le sentiment- et nous l'avons beaucoup entendu dire lors des auditions que nous avons réalisées -que si la création de cet établissement n'aboutit pas avec cette proposition de loi, il ne verra jamais le jour. En d'autres termes, c'est maintenant ou jamais raison pour laquelle il me paraît essentiel de ne pas trahir la confiance que votre personnalité a permis de rétablir. En effet, les deux défis auxquels la filière musicale, dans son ensemble, est confrontée, rendent nécessaire la création d'un établissement pour mieux y répondre et favorisent en même temps le regroupement de cette filière. Le premier défi est celui de la révolution numérique. Parmi les industries culturelles, la musique est le premier secteur à avoir été frappé par la crise due à l'arrivée d'innovations numériques révolutionnant la consommation de produits culturels. Un secteur autrefois florissant a ainsi été très brutalement confronté à une perte massive et rapide de revenus. L'édition phonographique est cependant parvenue à renouveler son modèle économique et ses modes de production pour renouer avec la croissance, comme le relève notre collègue Françoise Laborde dans son rapport pour avis sur le dernier projet de loi de finances, qui a souligné que, depuis 2013, le chiffre d'affaires du avait été multiplié par près de trois et le nombre d'écoutes par Cette crise contraste avec la situation, comparativement bien meilleure, du spectacle vivant, qui représente maintenant presque le double du poids de la musique enregistrée. Les concerts sont en quelque sorte devenus un nouvel eldorado pour l'industrie musicale, même si cela ne va pas sans un certain nombre de difficultés, à une concentration croissante des acteurs et au poids du financement de la sécurité. Je vous renvoie aux nombreuses communications faites à ce sujet, ces deux dernières années, par notre collègue Sylvie Robert, rapporteur pour avis des crédits du

secteur subventionné et secteur privé, musique « savante » et musiques populaires, pratique professionnelle et pratique amateur ... Les différents acteurs n'ont, jusqu'à présent, pas su construire une culture commune et présenter un front uni pour défendre des intérêts communs et valoriser le secteur. Devant ce constat, la proposition de loi prévoit la création, au 1 janvier prochain, d'un établissement public à caractère industriel et commercial, un ÉPIC, placé sous la tutelle du ministère de la culture et dénommé « Centre national de la musique La commission de la culture a adopté, il y a deux semaines, plusieurs modifications au texte que l'Assemblée nationale nous avait transmis pour clarifier et conforter les missions du futur établissement et mieux reconnaître la place des collectivités territoriales dans la définition et la mise en oeuvre de la politique de la musique. Pouvons-nous pour autant dire que le travail est achevé avec le texte de cette proposition de loi ? Comme le disait Miles Davis, « la véritable musique est le silence et toutes les notes ne font qu'encadrer ce silence Or, monsieur le ministre, il y a dans ce texte deux silences et, comme souvent avec les silences, ils concentrent toute l'attention. Un premier silence concerne la gouvernance du nouvel établissement. La composition du conseil d'administration d'un ÉPIC relève du pouvoir réglementaire. Le Parlement n'a donc pas véritablement la main sur les modalités de sa gouvernance. Or nous avons précisément constaté que ces questions de gouvernance font partie de celles qui agitent particulièrement la filière musicale, pour ne pas dire qu'elles la divisent ! Il ne faudrait pas que le projet achoppe sur ces questions, au motif que les solutions retenues, comme aurait pu le dire le regretté Michel Berger, dressent les acteurs « les uns contre les autres », alors que l'objectif est au contraire de faire en sorte qu'ils travaillent les uns avec les autres ! Il me paraît essentiel que les différents acteurs de la filière musicale n'aient pas le sentiment d'y perdre en se rassemblant au sein de cette nouvelle maison commune, faute de quoi le risque serait que certaines des associations de droit privé refusent de rejoindre le CNM, ce qui ferait perdre beaucoup de son intérêt au projet.

Je voudrais pour ma part souligner que les collectivités territoriales, chères au Sénat, ne doivent pas être les oubliées de cette gouvernance, au regard de leur contribution à l'animation et au financement de la politique musicale dans les territoires. second silence, c'est plutôt, de Pink Floyd, qui illustrerait parfaitement la situation ... La question des moyens du CNM est en effet au coeur de toutes les préoccupations. En l'état actuel, le CNM devrait percevoir la taxe fiscale sur les spectacles de variétés, des subventions de l'État et des fonds accordés volontairement par les organismes de gestion collective. Il devrait également gérer deux crédits d'impôt, soit un budget total de 78 millions d'euros.

Je vais vous poser la question le plus directement possible, monsieur le ministre : quels moyens supplémentaires vous est-il permis d'espérer dans le cadre du projet de loi de finances ? De votre réponse, même partielle, dépend beaucoup le sort du CNM, qui sera lié à la confiance et à l'engagement des acteurs, privés comme publics.

ces dernières années. Notre présidente, Catherine Morin-Desailly, avait émis l'idée d'affecter la taxe dite « YouTube » au bénéfice de la musique, qui est tout autant piratée que le cinéma.

Par ailleurs, le CNM aura-t-il les moyens de financer le fonds de soutien aux créateurs musicaux, envisagé à hauteur de 5 millions d'euros et dont la mise en place, je peux vous l'affirmer, est ardemment souhaitée par la profession, tant l'acte de création est absolument essentiel

J'estime pour ma part que votre soutien à la proposition de loi constitue un engagement moral qui doit trouver sa concrétisation dans le prochain projet de loi de finances. Ces silences, monsieur le ministre, il faudra bien les orchestrer afin d'éviter la cacophonie d'une filière une nouvelle fois déçue et trahie dans ses attentes. Or, tant que ni les structures de gouvernance ni les moyens ne sont arrêtés, ce sont plutôt des divisions qui sont créées, alors même que l'unité- vous l'avez dit -devrait prévaloir. Pour conclure, permettez-moi d'évoquer ceux qui sont au centre de l'ensemble de l'écosystème de la musique en France et que le Président de la République lui-même a salués comme il se doit au moment du débat sur la directive Droit d'auteur dans le marché européen : je veux parler des auteurs-compositeurs. Les industries culturelles reposent sur l'existence d'oeuvres. Leur prospérité dépend donc directement de la phase initiale de la création, qui implique l'intervention des auteurs-compositeurs.

Après huit ans de réflexion, nous ne pouvons donc que nous réjouir de la création d'une maison commune de la musique. Cette maison commune va devoir répondre aux attentes de la filière, être un outil efficace, une instance de dialogue et de cohésion entre les acteurs du secteur de la musique et des variétés.

Pour rester dans le jeu, nous devons renforcer les moyens financiers, mais également progresser en matière de compréhension et de capacité d'anticipation, condition pour faire face à la concurrence d'autres pays, en particulier les États-Unis et la Chine. Le CNM doit répondre à la volonté déterminée de maintenir la création et la production françaises dans une énergie et une vitalité qui permettent à chacun des acteurs d'en vivre, et ce sur tous nos territoires. Ces moyens sont autant un soutien financier qu'un soutien à la structuration et au développement par du conseil et de l'expertise fondés sur une observation la plus fine possible de l'écosystème, anticipant ses transformations itératives. N'oublions pas que la musique est une industrie culturelle qui pèse et représente de très nombreux emplois ailleurs que dans les métropoles. Au moment où la fracture territoriale est reconnue comme un problème central, ce point a toute son importance. Quatre grands enjeux doivent être au coeur des missions du CNM. Il s'agit en premier lieu de garantir la diversité musicale et le pluralisme des genres musicaux : tous les genres musicaux doivent avoir leur place au sein du CNM. Une attention particulière devra être portée à la musique classique et aux musiques improprement appelées « savantes ». « savantes ». Le financement des orchestres et des conservatoires, en région notamment, doit donc être conforté. Ceux-ci sont partout sur le terrain des vecteurs importants d'une grande part de la culture musicale. Ils n'ont pas le poids économique de formations et de groupes plus populaires, mais ils occupent néanmoins une place essentielle. Au coeur du CNM figurera aussi le répertoire historique du CNV : les musiques actuelles, le jazz et la variété, y compris l'humour. Parce que le CNM est un établissement public au service de l'intérêt général, il aura pour mission de garantir la diversité dans toutes les dimensions du secteur musical.

La diversité prend en compte les contributions de tous les acteurs, professionnels ou non, participant à la vie musicale en tant que créateurs, producteurs, diffuseurs, praticiens, spectateurs, auditeurs. La pratique musicale en amateur contribue aussi au développement de l'art musical français, à l'économie musicale et même au dynamisme des territoires. Mais cette vitalité tient également à la dynamique associative musicale.

promouvoir la diversité de la production et de la création musicales dans le monde, par le rayonnement français. La contribution française doit être accompagnée, aidée, encouragée. Il importe de favoriser le développement d'oeuvres françaises et francophones éclectiques à travers le monde. export de la musique française : à l'heure où l'exposition internationale des artistes et des productions français est une question cruciale pour la filière, cela permettra sans doute d'être plus efficace en matière d'export. La promotion de la chanson francophone est nécessaire. Nous la devons au monde, auquel la langue française apporte des valeurs et des façons de penser différentes, singulières.

La fusion en une seule et unique instance ne doit pas être synonyme de concentration : la concentration, c'est la négation de la diversité. Les inégalités culturelles sont nombreuses, trop nombreuses en France. Qu'ils vivent en milieu rural, insulaire, montagnard, ultramarin ou urbain, nos concitoyens doivent avoir accès à la culture.

Premièrement, de la gouvernance de l'établissement ? Les modalités devraient en être déterminées par voie réglementaire. Je souhaite insister sur l'importance du rôle des collectivités territoriales, qui participent de façon majeure à la politique publique de soutien à la musique, notamment le financement ou le subventionnement d'orchestres, de théâtres, de festivals, de conservatoires, d'écoles ou

prochain projet de loi de finances, et en particulier la question de l'administration des crédits d'impôt en faveur de la production phonographique et du spectacle vivant. Nous nous interrogeons

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la création tant attendue du Centre national de la musique témoigne de la volonté des parlementaires et du Gouvernement de mettre la filière musicale sur le devant de la scène de nos politiques culturelles. En dotant la France d'une maison commune dédiée à ses artistes, auteurs, compositeurs et interprètes, en unifiant l'ensemble des acteurs du monde de la musique,

qui concrétisera dès janvier 2020 ce projet mûri de longue date par vous-même, monsieur le ministre. Sont dessinés les contours de la future institution qui fera rayonner la musique française dans nos villes, dans nos campagnes, sur les plus grandes scènes internationales.

La proposition de loi reprend les grandes lignes du rapport des députés Pascal Bois et Émilie Cariou. Le Gouvernement n'a pas souhaité préciser, à ce stade, la gouvernance du CNM.

aux fonctions de direction, entre les femmes et les hommes, et n'est en rien épargné par les comportements sexistes. Nous appelons le Gouvernement à exercer la plus grande vigilance et à proposer des mesures fortes pour lutter contre la culture du sexisme qui gangrène l'ensemble de ce secteur.

Il s'agit de donner au futur centre les moyens de ses ambitions en résolvant une difficile équation : octroyer à la filière des ressources nouvelles et pérennes sans pour autant creuser le déficit public. ces besoins de financement sont d'autant plus importants, notamment pour les entreprises musicales, que le secteur s'engage depuis une dizaine d'années dans une profonde mutation. Les opportunités de développement à l'international sont décuplées avec le virage numérique. Nous devons accompagner au mieux les entreprises musicales françaises dans leur renouveau en consolidant leur modèle économique, afin de nous inscrire parmi les leaders mondiaux nous inscrire parmi les leaders mondiaux en matière de productions culturelles. Le Centre national de la musique a aussi une vocation de développement territorial de la filière musicale, en partenariat avec les collectivités locales, comme l'a réaffirmé la commission de la culture du Sénat.

-qui maillent notre territoire versent plus de 80 % des subventions dont bénéficient les lieux de musiques actuelles. Il nous semble essentiel, monsieur le ministre, de faire du Centre national de la musique un élément structurant du développement territorial de la filière musicale.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, sans revêtir les habits du thuriféraire et en restant comme toujours parfaitement objectif, je tiens, monsieur le ministre, à saluer ici la persévérance qui a toujours été la vôtre sur ce dossier. En avril 2011, le ministre de la culture de l'époque, un de vos nombreux, trop nombreux, prédécesseurs, vous confiait la conduite d'un rapport ministériel sur l'état de la création et de la diversité musicales à l'ère numérique. Huit mois plus tard, en novembre 2011, vous et vos quatre corédacteurs remettiez à Frédéric Mitterrand un document dressant, sans détour ni fioritures, le triste bilan économique et social de l'industrie française du disque entre 2000 et 2010. Avec Alain Chamfort, Daniel Colling, Marc Thonon et Didier Selles, vous proposiez notamment la création d'un centre national de la musique, sur le modèle du Centre national du cinéma, afin de sortir la filière musicale française du marasme qu'elle traversait et qu'elle continue de traverser. Huit ans plus tard, c'est avec une autre casquette, celle de ministre de la culture, que vous êtes parvenu à faire que ce centre puisse- enfin ! -devenir réalité, à l'horizon très proche de janvier prochain huit années pour arriver à mettre en oeuvre ce qui apparaissait comme une nécessité autant que comme une évidence. Bien sûr, les changements politiques de 2012 et les effets prolongés de la crise de 2008 expliquent pour partie que, alors qu'il convenait qu'il convenait d'agir vite, nous avons au contraire adopté l'attitude et la vélocité de l'escargot. En effet, entre 2012 et 2017, le budget dédié au ministère de la culture a diminué graduellement, avant d'afficher un léger sursaut, à la fin du quinquennat, pour contenter quelque peu la filière la filière musicale à l'approche des grandes échéances électorales. Mais, au-delà de la question strictement budgétaire, c'est l'absence de volontarisme politique dans le domaine de la culture durant tout un quinquennat qui explique sans doute le mieux ce retard à l'allumage. Entre l'annonce de sa création, fin 2011, l'arrêt du projet, en septembre 2012, l'annonce de sa relance, en janvier 2014, puis son nouvel arrêt, et enfin sa énième relance, en avril 2018,

a subi de coupes jusqu'en 2016, et combien de moyens il a fallu dégager depuis lors pour lui redonner un peu du lustre qu'il mérite une pratique, monsieur le ministre, qui honore le gouvernement que vous servez, notamment sur les questions culturelles, et s'agissant en particulier de la création du CNM, c'est précisément que vous vous attachez à tenir les promesses de vos prédécesseurs plutôt que d'en faire de nouvelles, avec l'arrière-pensée de les laisser à la charge d'éventuels successeurs ! En politique, je suis, comme vous, monsieur le ministre, de ceux qui pensent que la démagogie et les promesses non tenues sont le meilleur terreau sur lequel prospèrent les pires des populismes. C'est aussi, sans doute, votre implication personnelle, profonde et quasiment historique sur ce dossier qui explique que vous ayez réussi le tour de force de faire adopter ce texte à l'unanimité par l'Assemblée nationale, le 6 mai dernier. Néanmoins, mes collègues ayant déposé un nombre non négligeable d'amendements, vous devrez certainement patienter encore un peu avant que le texte soit définitivement adopté. Je veux toutefois souligner ici que, grâce au travail de très grande qualité conduit par notre rapporteur et à sa louable capacité de persuasion, seul un nombre restreint d'amendements ont reçu l'approbation de notre commission ce matin.

L'enjeu, on le sait, est de taille ; c'est pourquoi je suis persuadé que vous ferez tout, monsieur le ministre, pour répondre à l'inquiétude des professionnels du secteur, qui réclament que le futur Centre national de la musique soit doté d'un budget supérieur à celui des entités qu'il va regrouper en son sein. Nous souhaitons tous que le CNM montre au plus vite son utilité et son efficacité, comme l'a fait son lointain cousin, le Centre national du cinéma. Créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce dernier a su rapidement faire ses preuves ; il apparaît aujourd'hui comme une référence internationale en matière de politique culturelle sectorielle efficiente. On attribue souvent à Platon les mots suivants : « si l'on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique ». Dans un registre un peu différent, le cinéaste Alain Resnais déclarait en 1997, à l'occasion de la sortie de son superbe film intitulé, que « les chansons constituent les chansons constituent la mémoire historique affective de la France ». Oui, la musique et la chanson sont les coeurs sensibles et battants de notre culture. Elles appartiennent à notre patrimoine et sont un incroyable foyer de création artistique ; elles sont aussi un formidable vecteur de transmission et de démocratisation des savoirs. À ce titre, elles méritent pleinement que l'on crée un centre national qui leur soit entièrement dédié. Monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que le groupe La République En Marche votera en faveur de l'adoption je vous remercie Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, en l'an 303 avant notre ère, Cnæus Flavius, devenu édile curule à la suite d'un conflit avec les patriciens, fit construire un temple à Concordia, sur le Comitium, à Rome. Cette déesse était issue de deux divinités grecques,, dont le nom évoquait la sympathie des coeurs, et, qui présidait à la cohésion sociale et aux rapports harmonieux entre les citoyens et dont on tira un mot évoquant l'association heureuse de plusieurs sons. Ainsi, Concordia protégeait à la fois l'accord des coeurs et l'accord des cordes. Mais, pour réaliser son projet, Cnæus Flavius ne put obtenir d'argent public et se contenta du fruit des amendes imposées aux usuriers. Nous verrons dans la suite de la discussion, monsieur le ministre, si vous n'avez pas agi de même C'est sous les auspices favorables de cette même Concordia que le nouveau Centre national de la musique voit le jour, tant cette « maison commune de la musique » était attendue par toute la profession pour renforcer ses capacités d'action, pour s'adapter aux nouvelles modalités d'écoute et pour continuer de développer les pratiques, dans dans la richesse de leur diversité. L'État participe à la construction de cette nouvelle arche pour soutenir la filière, les créateurs, le rayonnement international de leurs oeuvres, mais aussi parce qu'il souhaite confier à ce nouvel établissement un rôle majeur pour déployer les politiques publiques du ministère de la culture dans les territoires. Je n'apporterai pas de voix discordante à ce concert de bonnes intentions. Indubitablement, il était nécessaire de rationaliser et de renforcer les moyens d'intervention des structures existantes, afin de mieux défendre l'exception culturelle française et de déployer l'égalité des droits culturels dans tous les territoires. Néanmoins, monsieur le ministre, nous attendons de ce débat qu'il éclaire davantage les projets politiques et les engagements budgétaires par lesquels votre ministère compte accompagner la création et le développement de ce nouveau centre. Dans son rapport, notre collègue député Pascal Bois, auteur de la présente proposition de loi, considère que la constitution du Centre national de la musique sera l'occasion, pour le Gouvernement, « de se doter d'une stratégie de long terme pour la politique publique de la musique, qui constitue l'une des missions fondamentales du ministère chargé de la culture ». Peut-être le dépôt d'un projet de loi par votre ministère aurait-il été plus approprié pour atteindre cet objectif. Alors que votre collègue le ministre de l'action et des comptes publics vient d'achever sa tournée des ministères afin de leur demander de réduire leurs budgets pour l'année 2020, nous nous interrogeons sur la capacité de votre ministère à participer au fonctionnement du futur centre national. De l'avis unanime, un apport de 20 millions d'euros est indispensable pour rassurer les membres constitutifs de la future entité et persuader tous les acteurs de la filière

nous souhaiterions que vous nous précisiez quelles politiques publiques, dans le domaine de la musique, vos administrations centrales continueront à gérer, et avec quels moyens. La semaine dernière, le Sénat a exprimé ses plus grandes réserves sur la création d'une Agence nationale du sport, qui aura sans doute pour conséquence la disparition du ministère de tutelle. tutelle. À ce propos, je citerai le jugement de Jean-Marc Sauvé, grand commis de l'État et secrétaire général du Gouvernement de quatre Premiers ministres successifs : « Depuis une quarantaine d'années, l'État s'est affaibli, moins par le transfert de compétences vers l'Union européenne ou vers les collectivités territoriales que par la réduction de ses capacités et de ses ressources en matière de conception et de stratégie. Aujourd'hui, la situation est telle que les grands opérateurs de l'État sont devenus plus puissants et plus experts que les directions des ministères chargées d'exercer leur tutelle. [ ...] L'" agencification " de l'État est aussi un facteur d'affaiblissement des services territoriaux de ce dernier. » Nos craintes portent aussi sur le financement du Centre national de la musique. Nonobstant vos réponses sur le montant de la subvention de l'État, ce financement sera constitué par l'agglomération de dispositifs déjà existants la taxe sur les spectacles vivants, pour une large part, les contributions des organismes de gestion collective, dans des proportions qui dépendront de leur implication dans la nouvelle structure, et les crédits d'impôts dont elle recevra la gestion en vue de développer des politiques incitatives.

Je rappelle que la Commission européenne considère le crédit d'impôt comme une aide d'État compatible avec les règles de la concurrence à la condition expresse qu'il favorise l'émergence de nouveaux talents. en ce qui concerne la taxe sur les spectacles, j'aimerais joindre, en parfaite harmonie, ma voix à celle de notre rapporteur, dont je salue la qualité du travail, pour souligner qu'il s'agit d'une taxe affectée, collectée sur une assiette restreinte, qui devra financer des dépenses beaucoup

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà quelques années, une émission diffusée par le service public annonçait que c'était « Ce soir ou jamais Pour le Centre national de la musique, c'est maintenant ou jamais ! Tout à fait ! En effet, une décennie après les premières ébauches de cette maison commune de la musique, il est enfin temps que le projet se concrétise.

les acteurs de la filière, qui se connaissent pourtant parfaitement, n'ont guère de lieux où échanger, partager leurs analyses du secteur, réfléchir collectivement aux mutations constantes qui le traversent. En somme, ils ont besoin de pouvoir se rassembler, dans leur diversité. Le futur CNM doit être ce lieu de rassemblement. Si cette assertion paraît simple, elle n'en recouvre pas moins une grande ambition, car réunir producteurs, éditeurs, diffuseurs, distributeurs, organismes de gestion collective et, bien entendu, artistes du privé ou du public, oeuvrant

À cet instant, je voudrais saluer l'esprit qui anime l'ensemble des acteurs de la filière, qui ont su, ces dernières années, faire des pas les uns vers les autres. Ils attendent aujourd'hui avec beaucoup d'impatience la création du CNM. L'instance de préfiguration animée par Catherine Ruggeri continue d'y contribuer. Ce périmètre élargi, où prévaut l'« égale dignité des répertoires », selon la belle expression de notre rapporteur, ne va pas sans soulever de véritables questions. À défaut d'avoir pu toutes les aborder par voie d'amendements- je pense par exemple à la question de l'aide à l'emploi -, le Parlement ayant encore été soumis, vous l'imaginez bien, à une interprétation pour le moins rigoureuse des articles 40 et 45 de la Constitution, je souhaiterais souligner, dans le cadre de cette discussion générale, plusieurs points qui me paraissent essentiels.

implique vraiment de changer de dimension. Plus précisément, il faut que cette nouvelle dimension soit en cohérence avec l'ambition désormais affichée. Pour le dire plus clairement, le CNM ne peut pas

doit plutôt être force de propositions à destination de la filière, mobilisateur sur les dossiers épineux du moment, stratège sur les grands enjeux. Tout en cultivant le dialogue et en coconstruisant avec les acteurs du secteur, il doit surtout être l'arbitre

Parce qu'il me paraît intéressant d'insister sur le caractère dynamique des missions revenant au CNM, je présenterai deux amendements visant l'un à inscrire dans le texte la mission prospective du futur centre national, l'autre à préciser que l'Observatoire de l'économie du secteur musical

dispositifs à instituer dans l'avenir. Au fondement de la chaîne de valeur de la filière musicale réside l'acte de création, et au fondement de la création artistique se trouve bien sûr l'artiste, le créateur de la valeur. Rendre l'artiste visible, c'est donner

... Monsieur le ministre, je crois que nous sommes unanimes, dans cet hémicycle, à ne vouloir à aucun prix que le CNM soit une coquille vide, une demeure hospitalière et prometteuse, mais vouée à l'abandon. Pour éviter ce funeste destin, il est impératif que les financements soient à la hauteur.

tous les musiciens se souviennent de la célèbre réplique d'André Malraux, interpellé à la Chambre sur l'absence de toute politique musicale d'envergure : « On ne m'a pas attendu pour ne rien faire pour la musique ! peut adhérer tout à fait à cette affirmation, car le directeur de la musique d'André Malraux, Marcel Landowsky, fut l'un des pères fondateurs de la politique musicale telle que nous la connaissons aujourd'hui, il semble temps de passer à une nouvelle phase dans le soutien à la musique, en lui donnant un centre national capable de rassembler, de renforcer et de représenter les intérêts de la filière, tout en soutenant ses exportations à l'international. je vous remercie de la constance de votre action en ce domaine et de la qualité des concertations menées par votre ministère avec l'ensemble de la filière musicale. Si la proposition de loi que nous étudions aujourd'hui est une étape nécessaire dans le parcours chaotique de la création du Centre national de la musique, elle n'apporte en réalité que peu de précisions sur le futur établissement public.

Il me semble en effet essentiel que l'État, qui est à l'initiative sur ce dossier, apporte une quote-part significative au fonctionnement du futur établissement public. Les financements innovants qui seront mobilisés nous intéressent au premier chef.

Il me semble normal que les poids lourds de la diffusion en ligne de contenus musicaux, compte tenu des bénéfices qu'ils en tirent, entrent dans le cercle vertueux du financement de la création musicale

à même de soutenir l'innovation et l'exportation, que nous appelons tous de nos voeux ! Bien qu'aucune politique publique ne puisse sérieusement se concevoir sans une connaissance et une observation fines du secteur, la musique reste l'une des rares filières à ne pas disposer d'observatoire. Alors que la loi LCAP avait déjà prévu la création d'un observatoire de l'économie de la musique au sein du CNV, certains blocages regrettables n'avaient pas pu être surmontés. Il est Il est strictement impossible de prétendre réguler un secteur sans s'appuyer sur des études précises, par exemple sur l'ampleur des phénomènes de concentration les et leur incidence sur la diversité. J'espère que le volontarisme dont vous faites preuve sur cette question permettra d'installer durablement un observatoire efficace, sans reproduire les erreurs passées. Comme je le soulignais dans mon rapport pour avis sur la mission « Médias, livres et industries culturelles » du projet de loi de finances pour 2019, la musique a été très tôt touchée par la révolution du numérique, mais elle a su y répondre rapidement et inventer un autre modèle durable, devant être encore consolidé. Les plateformes de diffusion de vidéos en ligne, si elles peuvent être porteuses de risques liés à la concentration tenant à l'usage d'algorithmes, constituent toutefois un moteur de croissance pour le secteur Il faudra sécuriser et préserver ce modèle de développement, qui est au coeur de l'avenir de l'industrie musicale. Aujourd'hui, dans le contexte d'une concurrence internationale impitoyable, nous devons conquérir de nouvelles parts de marchés à l'étranger tout en préservant la diversité musicale. C'est indispensable pour gagner la bataille des contenus, offrir à notre jeunesse des perspectives d'emploi durable, mais aussi donner à nos territoires de nouveaux atouts en matière d'attractivité. L'intégration du Burex, s'il y consent, au CNM, comme prévu à l'article 5 du projet de loi, participe de cette stratégie culturelle de conquête, à laquelle il faut donner la plus grande latitude. Cet acte de dissolution volontaire, qui concerne aussi les autres associations de droit privé ayant vocation à être intégrées au CNM, ne sera consenti que si un certain nombre de garanties sont apportées, permettant de présumer la puissance future du CNM. Il nous reviendra de veiller tout particulièrement au montant des subventions supplémentaires accordées au CNM par rapport aux subventions actuelles, car si l'une des associations venait à refuser l'intégration pour cause de financement insuffisant, c'est toute l'architecture du CNM qui serait fragilisée.

des amendements. Je confirme que le groupe du RDSE souhaite vivement faire advenir la création d'une maison commune pour la filière musicale, et ce dans les meilleures conditions possible. Nous attendons de nos débats une avancée sur la contribution financière de l'État et les taxes, ainsi que sur la composition des conseils,

grâce à vous- personne ne le conteste -et au député Pascal Bois, que vous avez encouragé à déposer cette proposition de loi pour mettre fin à cette douche écossaise

le théâtre, les arts de la rue et le cirque et, bien entendu, le cinéma. Il faut dire que vous y teniez, à ce Centre national de la musique ! Vous aviez autrefois émis un rapport très favorable à sa création. À la commission de la culture du Sénat, en phase avec vos propositions. D'entrée de jeu, nous exprimons notre satisfaction devant cette proposition de loi tant attendue. La musique étant une amie de la vie quotidienne de chacun de nous, on finit par oublier qu'elle n'existe que dans le cadre d'une vraie filière, certes culturelle, mais aussi économique et industrielle. Il était temps de structurer cette filière, d'autant que la révolution numérique a fait souffler sur elle la tempête que nous connaissons.

le Fonds pour la création musicale, le Burex, le Club action des labels et des disquaires indépendants et le Centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles. Ces derniers organismes pourront transférer leurs ressources au futur CNM et se fondre en lui dès qu'ils auront entériné leur dissolution,

Cette habilitation octroyée au président du CNM constitue une marque de confiance envers le nouveau centre national et lui confère d'emblée une certaine crédibilité auprès du secteur de la musique, en le positionnant comme un acteur incontournable.

Le rapprochement entre les OGC et le CNM est légitime et souhaitable. Le montant total de ces ressources s'est élevé, en 2017, à 183 millions d'euros, somme dont la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteurs et des droits voisins

de ce texte permettra de regrouper différentes structures publiques et privées au sein d'un seul et même établissement. À l'heure des mutualisations et des économies d'échelle, elle devrait donner un nouveau souffle à la politique musicale en France, qui est à la peine depuis une décennie, notamment sur la scène internationale. En effet, si la musique est omniprésente dans notre quotidien, le secteur est « en crise » depuis longtemps ; il mérite toute notre attention. C'est la deuxième industrie culturelle en France, derrière celle du livre ; elle est talonnée de près par le jeu vidéo. En France, la musique pèse 8,7 milliards d'euros, dont à peine 10 % pour la vente de musique enregistrée, et près de 240 000 emplois.

Oui, la musique est un art vivant ! Pourtant, c'est le seul qui ne dispose pas, à ce jour, d'un centre national. Si l'on peut se réjouir de la facilité avec laquelle la musique ponctue désormais notre quotidien, force est de constater que le piratage de masse-

au travers de ce texte devrait permettre de se doter d'une stratégie de long terme en matière de politique publique de la musique, de rassembler toute une filière- artistes, entreprises, organismes de gestion des droits d'auteur, etc. de créer un observatoire, de favoriser la création et la diversité, d'accompagner le développement de la production de la musique, de promouvoir l'innovation.

En effet, le conseil professionnel doit être élargi aux représentants des structures publiques de la musique en région, et il est important que la parité soit respectée au sein de cette instance.

le Centre national du cinéma et de l'image animée, ou CNC, doté de moyens significatifs et en mesure de faire dialoguer et coordonner les différentes composantes du secteur, il n'en va pas il n'en va pas de même pour la musique. En réalité, il s'agit du dernier art vivant qui ne dispose pas d'un centre national, au contraire de la danse, du livre, du théâtre, des arts de la rue, du cirque et, donc, du cinéma.

Création musicale et diversité à l'ère numérique », commandé par le ministre de la culture de l'époque, Frédéric Mitterrand. Écrit dans le contexte d'une industrie musicale largement en crise, notamment sous l'effet de la numérisation et du développement du, ce rapport préconisait la création d'un centre national de la musique. Comme vous le rappeliez, monsieur le ministre, quinze dernières années, l'industrie du disque a connu une crise de grande ampleur, notamment du fait du piratage de masse, avec une baisse de son chiffre d'affaires de l'ordre de 60 % entre 2002 et 2015.

d'une part sur la gouvernance de l'établissement, dont les modalités devraient être déterminées par voie réglementaire, d'autre part sur son financement, qui sera discuté lors de l'examen du prochain projet de loi de finances. Nous allons donc devoir nous prononcer sur la création d'une structure sans connaître son budget prévisionnel. Ces deux questions sur lesquelles les parlementaires votent à l'aveugle cristallisent les inquiétudes des acteurs. L'Alliance des entreprises de la musique, par exemple, qui regroupe les syndicats du spectacle vivant, de l'édition phonographique et de l'édition de musique, a apporté un soutien unanime au projet Toutefois, elle reste vigilante sur les questions budgétaires, puisqu'elle fait remarquer que les crédits d'impôt du spectacle vivant ont déjà été rabotés lors du vote de la dernière loi de finances. Il appartient au Gouvernement de confirmer son engagement de donner un souffle neuf à la politique musicale en assurant au nouvel établissement les moyens de remplir sa mission. La volonté de ceux qui ont imaginé le Centre national de la musique a été de ne pas « nationaliser » les structures associatives qu'ils projettent d'intégrer à la nouvelle structure. Aussi la dissolution des associations doit-elle être décidée par ses membres. Si les professionnels n'avaient aucune garantie sur l'efficacité de la structure et décidaient de ce fait de changer d'avis, la fusion proposée pourrait ne pas avoir lieu. Restons donc vigilants. Il y a aussi, à l'heure du numérique, un véritable problème d'inégalité de répartition de la richesse créée entre producteurs et artistes. Selon l'Adami, la Société civile pour sur 9,99 euros d'abonnement mensuel au, seulement 46 centimes vont aux artistes, contre 4,57 euros aux producteurs et 1,96 euro à la plateforme. Il est inconcevable que, au titre du musical,

afin de préciser que le CNM contribue à la mise en oeuvre de la politique publique en faveur de la musique et de centrer ses missions sur les artistes, dont il faut défendre les droits. Sans eux, rien ne serait possible. Nous souhaitons également préciser le rôle important des partenaires que sont les collectivités territoriales, en conférant une base légale aux contrats de filière qui existent déjà dans le secteur des musiques actuelles et de variétés et en autorisant d'autres types de partenariat. Mes chers collègues, nous ne rappellerons en effet jamais assez la place essentielle occupée par les collectivités territoriales en matière de déploiement du service public de la culture en général, et de la musique en particulier. Je regrette que notre que notre proposition que le CNM puisse être compétent pour mettre en oeuvre et gérer les dispositifs d'aide à l'emploi des artistes du spectacle du secteur des musiques actuelles ait été déclarée

La création du CNM nous offre donc une formidable occasion d'accompagner les investissements des entreprises de la musique sur un marché mondial en pleine expansion. Cet accompagnement doit être le coeur du réacteur du futur établissement, au service des projets des artistes et des auteurs, au service du rayonnement de la France et de la langue française partout dans le monde, au service des jeunes générations, auxquelles la filière va pouvoir proposer de nouveaux viviers d'emplois. Si cette stratégie de conquête a besoin d'être soutenue, cela tient aux spécificités du secteur. La prise de risque est le dénominateur commun à toutes les entreprises de la musique en ce qu'elles opèrent dans des industries dites de prototype, ce qui les conduit à un niveau très significatif de réinvestissement de leurs revenus dans la découverte de nouveaux talents en France. S'agissant de la musique enregistrée, l'an passé, sur les vingt meilleures ventes d'albums en France, dix-neuf étaient des productions françaises. Ce résultat doit beaucoup au talent de nos artistes et au travail de leurs labels, mais aussi, il faut le rappeler, au crédit d'impôt phonographique. Il faut se réjouir de l'efficacité de ce dispositif fiscal, défendu par le Sénat lors de l'élaboration de la dernière loi de finances, mais il faut aller plus loin, pour permettre aux artistes produits en France de se hisser parmi les meilleures ventes mondiales.

à la démocratisation de la culture, à la liberté de la création et de la programmation et à l'équité territoriale, permettant la coopération entre tous les acteurs. Il existe donc un réel risque de fragilisation et de démantèlement du ministère de la culture par le transfert de missions essentielles de la politique publique au Centre national de la musique. C'est pourquoi il est indispensable que le projet du CNM ne puisse entrer en concurrence avec les missions de service public du ministère

à l'État en matière de politique musicale. C'est pour cette raison que nous avons, par exemple, précisé que la politique en matière d'éducation artistique et culturelle relève de l'État et des collectivités et que l'Assemblée nationale avait déjà inscrit dans le texte le rôle clé joué par le ministère de la culture en matière de soutien au secteur de la musique et des variétés. La commission est défavorable

à resserrer le périmètre de cet alinéa, qui porte sur l'ensemble du secteur professionnel, en évoquant particulièrement le sort des artistes. L'alinéa suivant, en revanche, porte sur les différentes activités de la filière musicale. J'ai déposé un amendement qui devrait vous satisfaire, puisqu'il vise à préciser la notion de création afin de garantir un soutien aux auteurs, aux compositeurs et aux interprètes. C'est pourquoi je vous invite à retirer votre amendement, ma chère collègue. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

aux pratiques et aux composantes du secteur professionnel de la musique, j'estime que le CNM doit pouvoir garantir la diversité culturelle et la protection des droits de tous les acteurs du secteur, professionnels ou non. ou non. Cet amendement vise à couvrir un champ plus large que celui de l'alinéa 3, en étendant la garantie de la diversité musicale à tous les acteurs du secteur de la musique. Il s'agit de garantir le droit de tous à participer à la vie musicale de protéger les personnes contre le risque de censure, de contrôle injustifié des ressources musicales et de restriction des libertés. Quel est l'avis de

que vous souhaitez lui confier me paraît être davantage du ressort de l'État. D'ailleurs, j'observe que l'article 3 de la loi LCAP a donné pour objectif à la politique de la création de « garantir la diversité de la création et des expressions culturelles

il s'agit ici de donner toute la place qui leur revient aux auteurs, sans lesquels la musique n'existerait pas. Il me paraît primordial qu'ils soient mentionnés d'une manière ou d'une autre dans le texte, afin de reconnaître la place centrale qu'ils occupent au sein de la filière musicale. musicale. Cette filière s'appuie sur une multitude d'acteurs interdépendants, même si l'apparition de stratégies « à 360 degrés » depuis la crise du disque entraîne peu à peu une réduction de leur nombre. Quoi qu'il en soit, Quoi qu'il en soit, reconnaissons que c'est bien le talent et la créativité des auteurs, des compositeurs comme des artistes-interprètes qui en constituent le socle. Quelles que soient les évolutions qui sont intervenues ou qui interviendront encore dans le domaine de la musique, leur rôle reste aussi déterminant qu'irremplaçable. Nous avons mené une importante concertation avec toutes les parties prenantes. Je remercie spécialement le ministère de son aide. Nous sommes parvenus à une

bien ! Quel est l'avis du Gouvernement ?

ne constitue pas un métier de la musique et des variétés au même titre que la création, la production, l'édition, la promotion, la distribution ou la diffusion. Par ailleurs, la formation professionnelle constitue déjà l'une des missions dont devrait être chargé le nouvel établissement public, en application de l'alinéa

j'insiste sur ce point -et, éventuellement, de développer des offres de formation à destination des professionnels et des porteurs de projet du secteur, dans les cas où une carence de l'initiative privée aurait été identifiée. La commission est défavorable à cet amendement.

à l'oeuvre et mieux accompagner le secteur dans ses évolutions. Pour moi, cette mission de prospective doit irriguer l'action du CNM dans ses différentes directions,

Mme Françoise Laborde. Dans le secteur des musiques actuelles, la formation professionnelle n'est pas encore tout à fait structurée. Elle est assurée par des organismes de formation et des structures diverses, dont la formation ne constitue pas exactement le coeur de métier. Afin de soutenir la structuration de la future mission de formation du CNM et de pouvoir proposer une offre répondant aux réels besoins du terrain, il semble essentiel de s'appuyer sur une action de prospective, d'innovation et de développement des compétences

et peut-être avant tout, un travail de structuration de l'offre, pour garantir que celle-ci réponde aux besoins particuliers du secteur, notamment lorsqu'apparaissent des demandes de nouvelles compétences. La commission a donc émis un avis favorable

En prenant en compte l'évolution des usages au-delà des seules mutations technologiques, le CNM devrait être mieux à même d'accompagner le secteur et de proposer des aides plus ciblées pour remédier aux différentes difficultés auxquelles celui-ci est confronté.

Le CNM ne sera efficace que si cette union est réelle. Pour l'instant, les lieux de concertation et de dialogue manquent dans le secteur de la musique. On constate notamment une méconnaissance entre les acteurs et représentants de la musique enregistrée, d'une part, et ceux du spectacle vivant, de l'autre, alors que, bien souvent, ces activités sont liées. Le CNM doit être le point de convergence de toutes les discussions techniques et des actions conjointes autour de la musique.

les collectivités d'outre-mer sont déjà incluses à part entière dans le champ de la disposition. Au contraire, en mentionnant spécifiquement les collectivités d'outre-mer, ne donnerait-on pas le sentiment que, chaque fois que nous mentionnons les collectivités dans un texte de loi sans faire référence aux collectivités d'outre-mer,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

elle doit être construite et mise en oeuvre avec les collectivités territoriales. Cette mission de développement territorial du CNM permettra un effet de levier, en facilitant la mobilisation des collectivités au bénéfice des acteurs musicaux, gage d'un développement économique durable du secteur

avec les collectivités territoriales, les services déconcentrés de l'État et les différents acteurs professionnels et non professionnels de la filière musicale. Je le rappelle, ces contrats de filière ont déjà cours depuis 2017 dans le secteur des musiques actuelles et des variétés. Ils offrent un cadre commun pour la mise en oeuvre, dans un délai limité, de mesures nouvelles portées et financées conjointement, qui s'ajoutent, sans s'y substituer, aux dispositifs existants.

par des opérateurs bretons autour de cinq axes : accompagner des parcours de développement artistique ; aider au développement stratégique des entreprises de production encourager la collaboration entre les acteurs des musiques actuelles et des variétés ; développer les pratiques de coproduction des salles de musiques actuelles ; développer le numérique et les nouveaux usages. Cette formule existe et fonctionne également les régions Pays de la Loire, Normandie ou Nouvelle-Aquitaine, et il me semble important de lui donner une base légale. Par ailleurs, le CNM est appelé à fédérer l'ensemble de la filière, et je ne suis pas partisane d'exclure les non-professionnels de son champ d'action.

prévoit que le CNM participe au développement de l'éducation artistique et culturelle, en complément du rôle joué par l'État en la matière. L'éducation nationale étant concernée, il faut, en cohérence avec l'alinéa 14, préciser, à l'alinéa 15, que, parmi les entités avec lesquelles le CNM pourra

en tête -et par les collectivités territoriales. Il n'est pas souhaitable de lui octroyer la possibilité de conclure directement des partenariats avec les établissements scolaires en se substituant à l'action de l'État et des collectivités territoriales en ce domaine.

Inadaptée à l'histoire, à l'organisation et aux logiques économiques du secteur, la piste d'une grande " agence de la musique " paraît d'emblée devoir être écartée. L'heure n'est pas à la création, pour la musique, d'un équivalent du Centre national du cinéma et de l'image animée Une telle orientation, d'une part, se heurterait immanquablement et légitimement à de larges et fortes oppositions et, d'autre part, réduirait à néant les outils dont dispose l'État, en particulier au niveau au niveau déconcentré. Seule la mise en oeuvre de certains aspects de la politique musicale paraît susceptible d'être confiée à un opérateur. [ ...] À l'avenir, ces À l'avenir, ces administrations [centrales] et leurs relais déconcentrés devraient demeurer le lieu du soutien- direct et pérenne -aux structures qui reposent nécessairement sur la subvention publique. » On comprend bien que

Les règles de gouvernance doivent notamment permettre de garantir l'intérêt général dans un secteur où les intérêts particuliers des différentes parties prenantes ont parfois pris le dessus, de telle sorte que sont apparues des situations de conflit d'intérêts.

Si la détermination exacte du nombre de membres du conseil d'administration, de sa composition et de son fonctionnement peut relever du pouvoir réglementaire, la mention des principales catégories de représentants amenés à y siéger peut aussi relever du niveau législatif. C'est le choix

Il paraît nécessaire de garantir, en sus de celle de l'État, une représentation forte des collectivités territoriales,

La composition proposée par les auteurs de l'amendement n° 27 rectifié est un peu plus large, puisqu'elle comprend des représentants des professionnels du domaine de la musique et des variétés, sous forme enregistrée et de spectacle vivant, des représentants des OGC et d'autres personnalités qualifiées. Comme je l'ai indiqué en commission, je comprends parfaitement que la question de la gouvernance préoccupe tout le monde. Elle est absolument majeure pour la réussite de la création du CNM.

relève du pouvoir réglementaire. La loi prévoit que la représentativité des organisations syndicales s'apprécie à l'aune de différents critères, au nombre desquels figurent le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, l'ancienneté, l'audience, l'influence, ainsi que les effectifs d'adhérents et les cotisations. Ces critères ne sont cependant pas applicables à bon nombre d'organisations qui pourraient être appelées à siéger au sein du conseil professionnel. L'adoption de cet amendement contribuerait donc à créer une forme d'inégalité entre les organisations pouvant être concernées et les autres. Il me paraîtrait regrettable de tendre à exclure, par l'adoption du critère de représentativité, même modulé par l'emploi du terme « notamment », un certain nombre d'organisations de la possibilité de siéger au sein du conseil professionnel, alors que nous ignorons la manière dont sera composé le conseil d'administration. Il est important que les règles de gouvernance permettent

Je crois que nous en avons tous conscience ici. Cependant, je pense que nous devons nous en remettre au pouvoir réglementaire pour fixer la composition du conseil d'administration du CNM. La loi prévoit, par défaut, que les conseils d'administration des ÉPIC

Si tous ne peuvent être représentés au conseil d'administration ou au conseil professionnel, il nous semble légitime que des espaces, des plateformes de dialogue et de concertation puissent réunir l'ensemble des acteurs de la filière, ce qui constitue l'une des missions premières du CNM.

l'avis de la commission ? On ne peut qu'adhérer à l'esprit de cet amendement, qui définit ce que devrait être cette « maison commune » du Centre national de la musique. Cependant, la définition donnée, très générale, est plus du niveau du règlement,

sur les spectacles de variétés sera consacrée au financement du CNM. Cela soulève la question des bénéficiaires du produit de cette taxe. Il appartiendra au conseil d'administration de définir les entreprises éligibles,

C'est la condition du maintien d'un climat de confiance avec les entreprises de spectacle musical et de variétés. Nous souhaiterions, monsieur le ministre, avoir des précisions sur ce sujet.